que tous prennent leur retraite à cet âge. Cette dérogation concerne les métiers les plus pénibles : horaires atypiques, travail de nuit, mouvements répétitifs entraînant des troubles musculo-squelettiques. En réalité, moins de 5 % des salariés de la RATP

20 millions d'euros à 30 millions d'euros de cotisations retraite en moins chaque année. En raison de l'ouverture du marché à la concurrence, on estime qu'environ 19 000 salariés quitteront la RATP pour rejoindre des filiales ou des entreprises concurrentes. Cela entraînera inévitablement des difficultés de recrutement et des vacances de postes. La suppression de ce régime spécial aura donc des conséquences néfastes sur l'attractivité de la RATP. De même, dans le contexte actuel de bifurcation écologique, nous avons besoin de chauffeurs de bus et de métro, de techniciens, ainsi que d'ingénieurs de l'énergie. Nous devons donc reconnaître la pénibilité de ces métiers pour renforcer leur attractivité et pallier les difficultés de recrutement. Tel est l'objet de cet amendement.

et 2, qui ferment le régime spécial des retraites de la RATP. En effet, les salariés de la RATP sont soumis à des sujétions importantes et à une pénibilité particulière. Les conditions de travail se dégradent de plus en plus horaires atypiques, fréquence des astreintes, usure physique, mais aussi augmentation des incivilités auxquelles les agents sont confrontés ... Tout cela affecte la condition physique et mentale des travailleurs. S'y ajoute le recours, désormais systématique, au travail de nuit, afin d'augmenter la productivité, ce qui dégrade également les conditions de travail. Les conducteurs de bus, eux, sont confrontés à la dégradation continue des conditions de circulation sous l'effet de la densification de la population et des nouvelles mobilités,

la retraite. Les transports franciliens- le métro, le RER et le bus -subissent tous des sous-effectifs de conducteurs, ce qui a largement dégradé les conditions de transport au cours des derniers mois pour les habitants de la région parisienne. Comment recruter quand on réduit encore l'attractivité des métiers ? La parole

Les transports franciliens- métro, RER, bus -, en plus de devoir assumer la réorganisation totale due à l'ouverture à la concurrence, que notre groupe a combattue lors de l'examen de la loi d'orientation des mobilités en 2019, subissent une crise majeure de ressources humaines. Le mal-être des conducteurs, notamment des conducteurs de bus, est immense, comme le prouvent les mouvements sociaux, particulièrement en grande couronne. Dès lors, comment pallier les problèmes de recrutement si l'on réduit encore davantage l'attractivité des métiers ? Nous ne comprenons pas votre logique Le mouvement « Stop galère » a été lancé par les associations d'usagers et partis de gauche d'Île-de-France cet hiver face à cette triple ineptie : attaque sociale contre les travailleurs de la RATP, hausse du passe Navigo, baisse des financements. Ce n'est pas aux travailleurs et aux usagers de payer les pots cassés d'une mauvaise réforme des retraites et d'une mauvaise compensation par l'État des pertes de recettes d'Île-de-France Mobilités du fait de la crise sanitaire comme des mauvais calculs en vue du Grand Paris Express. Enfin, le Gouvernement et la majorité sénatoriale n'ont de cesse de crier à l'injustice contre la situation qui prévaut en Île-de-France et celle des autres réseaux de transports en commun dans le pays. Mais pourquoi toujours vouloir niveler les régimes par le bas ? Vous voulez supprimer le régime spécial de la RATP, comme une conséquence de l'ouverture à la concurrence que vous, majorité sénatoriale, avez votée. Vous étiez alors moins silencieux.

de la RATP. Les horaires atypiques, la fréquence des astreintes ou encore l'usure affectent les conditions physiques et mentales des travailleurs. Il est indispensable de prendre en compte divers critères de pénibilité.

La question des transports est sans doute le point clé de la réussite de ces jeux et sera déterminante pour l'image de la France à l'étranger.

En jetant le discrédit sur les agents de la RATP, qui seraient des privilégiés, et en fermant ce régime spécial à compter du 1 septembre prochain pour les nouvelles embauches, vous compliquez la tâche de Jean Castex pour mener à bien son recrutement. Je sais que l'ancien Premier ministre devient encombrant, surtout lorsqu'il visite avec bonhomie et succès le salon de l'agriculture, mais ce n'est pas une raison pour lui mettre des bâtons dans les roues. nous le savons, la fermeture du régime spécial des agents de la RATP, est au mieux un artifice, au pire un appât pour se concilier une soi-disant opinion publique et s'en octroyer les faveurs, de faire passer une réforme qui n'est en réalité que brutale et surtout pas nécessaire.

bus connaissent actuellement, et singulièrement depuis la crise de la pandémie du covid-19, des sous-effectifs de conducteurs qui ont amplement dégradé les conditions de transport ces derniers mois. Cette question n'est pas seulement celle de la protection des salariés ; c'est aussi celle des usagers de la région parisienne, en particulier ceux ceux de la grande couronne, que je côtoie personnellement chaque jour. Comment recruter quand on réduit encore l'attractivité des métiers ? C'est une véritable question.

de nos réglementations et de notre législation à des conditions particulières relève de l'exigence de notre travail de parlementaires. Nous ne pouvons pas être dans l'uniformisation. Il faut tenir compte des règles particulières et, en l'occurrence, ne pas faire disparaître ce régime spécial.

En effet, les conditions de travail n'ont guère changé au sein de la RATP : il y a toujours des horaires atypiques, de la fréquence d'astreinte, du travail de nuit et des amplitudes horaires de l'usure qui affectent les conditions physiques et mentales des travailleurs. Ce n'est pas un régime privilégié ; c'est juste une mesure de justice sociale. Ainsi, plutôt que de niveler les droits des salariés par le bas,

Or la réalité particulière de chacun, vécue par les salariés de la RATP, n'est pas celle d'un régime usurpé ou favorisé. C'est au contraire celui d'une compensation accordée pour une vie au travail particulièrement dure. C'était la règle du jeu. Par ailleurs, les transports franciliens-

du travail de nuit, des astreintes, de l'usure physique, des conditions de circulation de plus en plus difficiles en Île-de-France et du stress lié au comportement d'un certain nombre de clients,

Les métiers de la RATP souffrent d'un véritable manque d'attractivité, et les Franciliens en ressentent les conséquences quotidiennement. Il suffit de prendre les transports en commun pour se rendre compte de l'effet du manque de personnels sur les réseaux franciliens. L'année dernière, sur 1 500 postes de chauffeurs de bus qui manquaient, seulement ont été pourvus. S'attaquer au régime spécial de la RATP, c'est rendre encore moins attractifs ces métiers et, par conséquent, aggraver les difficultés que le réseau connaît déjà. En outre, le projet de suppression du régime spécial de la RATP est à contretemps et paradoxal. En effet, rendre attractifs les métiers de la RATP, c'est rendre attractifs les transports en commun pour les Franciliens. vous vous en prenez une fois de plus aux services publics de transports, alors même qu'ils sont la solution face au réchauffement climatique, dont les effets dévastateurs sont dès aujourd'hui palpables.

Au contraire, vous les en dégoûtez et tombez dans le piège de l'écologie punitive. Mes chers collègues, pour éviter un nivellement par le bas pour les employés de la RATP

la conduite de plus en plus stressante, sans parler des horaires atypiques ou encore des astreintes. Ces conditions de travail dégradées ont des conséquences sur les plans physique et psychique pour les travailleurs de la RATP. Doit-on pour autant considérer ces derniers comme des privilégiés ? Il est indispensable de prendre en compte divers critères de pénibilité : c'est là que résident l'équité

Il est indéniable que les transports publics et, d'une manière générale, les mobilités connaissent actuellement des mutations technologiques, des révolutions d'habitudes, d'usages et de besoins probablement inédites depuis l'avènement du chemin de fer.

qu'au lieu de niveler les droits des salariés par le bas en supprimant les régimes spéciaux, il faut permettre à l'ensemble des salariés exposés à la pénibilité de partir plus tôt à la retraite. Les transports franciliens- le métro, le RER et le bus -subissent tous des sous-effectifs de conducteurs, ce qui a largement dégradé les conditions de transport au cours des derniers mois pour les habitants de la région parisienne.

L'article 1, dont nous parlons depuis ce matin, n'en est qu'une illustration parmi d'autres. La suppression des régimes spéciaux témoigne parfaitement du manque d'empathie dont font preuve non seulement

Ce métier fait particulièrement mal au dos. Je vous invite à l'essayer ne serait-ce qu'une journée : vous verrez ! C'est le résultat d'une combinaison de facteurs, d'ailleurs bien détaillés, de risques biomécaniques causés par les vibrations et de facteurs de risque aigus liés au port de charges. Comme par hasard, ce sont là deux des quatre risques que vous avez supprimés du compte professionnel de prévention, mécanisme que nous avions introduit par nos précédentes réformes. Avec l'article 1, le Gouvernement pousse encore plus loin la brutalité de 2017. Demain, les nouveaux travailleurs des régimes spéciaux relèveront mécaniquement du droit commun, c'est-à-dire du régime général, qui ne compense la pénibilité que de manière très insuffisante ; c'est le moins que l'on puisse dire. Les chauffeurs de métro, les mineurs, qui ne voient que rarement la lumière du jour, les chauffeurs de bus parisiens qui se lèvent tôt parce qu'ils habitent en banlieue ; tous ces travailleurs qui subissent la dureté de leur

alors bien plus bavards. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à repousser l'entrée en vigueur de la fermeture du régime spécial de retraite de la RATP à une date déterminée par décret pris en Conseil d'État après concertation des organisations syndicales et patronales, au plus tard

Je n'évoquerai pas le caractère injuste et brutal de la suppression de ce régime spécial : je privilégierai une approche très pragmatique. Comme chacun sait, au regard des enjeux liés à la nécessité de décarboner notre société, le développement des transports publics est indispensable. Il s'agit de réduire l'utilisation de la voiture individuelle.

vise, lui aussi, à repousser l'entrée en vigueur de la fermeture du régime spécial de retraite de la RATP à une date déterminée par décret pris en Conseil d'État, toujours après concertation des organisations syndicales et patronales, au plus tard au 1 janvier 2040.

pour la retraite complémentaire, les salariés nouvellement embauchés dans les secteurs et les organismes concernés seront affiliés à l'Agirc-Arrco, organisme géré de façon paritaire par les organisations patronales et salariales,

les contester, puisque je n'ai entendu aucun de mes collègues dire que les métiers de la RATP n'étaient pas, pour une bonne part d'entre eux, Malheureusement, vous ne semblez pas nous entendre ... Aussi, nous vous proposons une forme de compromis pour garantir aux salariés actuels qu'ils pourront bien bénéficier d'un départ à la retraite anticipée s'ils le souhaitent.

Si vous supprimez dès 2023, par l'amendement de M. Retailleau, la possibilité de bénéficier de ce régime, alors- cela va de soi -bon nombre de ceux

Cela veut dire que la situation financière de la RATP demeure fragile ; ses marges de manoeuvre sont extrêmement limitées. Il est donc nécessaire de donner du temps

de la retraite de la RATP à une date déterminée par décret pris en Conseil d'État, après concertation des organisations syndicales et patronales au plus tard le 1 janvier 2031.

alors qu'elle sera confrontée à des échéances particulièrement importantes, que nous devons tous ensemble réussir ; je pense par exemple aux jeux Olympiques. Ensuite, le moment est malvenu,

vous qui la bloquez ! ... il faut que la concertation réussisse à convaincre les premiers concernés et que nous puissions obtenir leur adhésion. L'amendement

Il s'agit de modifier la date de la fermeture du régime spécial de retraite de la RATP,

et patronales, en l'occurrence le patron Castex. Il faut un décret en Conseil d'État. Pour ma part, je proposerai une date qui me paraît bien plus raisonnable et qui permet de conduire cette discussion ; celle du 1 janvier 2030. Cela ne me semble pas trop rapide et laisse le temps d'approfondir les conditions qui permettraient de conduire cette fermeture du régime spécial de retraites, fermeture que par ailleurs nous ne souhaitons pas, mais qui pourrait éventuellement être adoptée par notre assemblée. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un amendement de repli.

où les gens ont de plus en plus de mal à vivre, où les salaires stagnent et ne sont pas à la hauteur, où les classes moyennes, qui se paupérisent, s'ajoutent à celles qui sont déjà pauvres, et où il y a une forte tension. l'on vient nous dire, alors même que certains font des milliards d'euros de bénéfice à la faveur de la crise, qu'il faut absolument faire payer de deux ans de leur vie les plus démunis du pays

Pour cette raison, il ne faut absolument pas adopter cette mesure ... Il faut conclure. ... parce qu'elle est hors temps.

rencontre des difficultés majeures, il est juste de préserver l'attractivité de tels métiers et de prendre du recul quant à l'ouverture prochaine de la mise en concurrence prévue pour les bus en 2025, pour les tramways en 2029 et pour les RER en 2039. Cette ouverture à la concurrence aura des conséquences aussi bien sur la qualité que sur la fiabilité du régime. Il nous paraît donc indispensable de préserver le régime spécial de la RATP, d'où nos amendements de suppression. Mais comme vous les avez refusés, nous vous présentons cet amendement de repli. Vous savez pertinemment que, malgré des campagnes de recrutement régulières, la RATP peine à attirer des salariés. Rien d'étonnant ! L'abandon progressif du statut a un effet négatif sur l'attractivité de l'entreprise, où 75 % du personnel travaille avec des horaires atypiques

supprimer ce régime spécial ne fera que dégrader les conditions de travail, donc les conditions de transport de millions de voyageurs en Île-de-France. Votre mesure va entraîner une dégradation brutale des droits des nouveaux entrants. Alors même que vous vous vantez d'un dialogue social au sein des branches, la réalité est que vous passez outre les discussions qui ont ont permis l'obtention de ce droit grâce à des négociations de branches justement, et vous balayez d'un revers de la main un régime qui a pour vertu de prendre en compte la pénibilité spécifique de cette filière. Tel est le sens de

est pourtant évident : à partir du 1 septembre 2023, les nouveaux embauchés des entreprises bénéficiant d'un régime spécial seront affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), donc au régime général de l'assurance vieillesse. Cela implique mécaniquement

contre le travail des enfants et contre le sénateur Thénard, partisan du maintien des règles sociales les plus dures. Mes chers collègues, soyons tous Hugo et ne soyons pas Thénard

vous avez ouvert le secteur à la concurrence. Or les salariés qui sont transférés dans le privé perdront leur statut, mais garderont leur régime de retraite. J'espère que vous suivez ... Pas trop ! Vous souhaitez un référendum sur les régimes spéciaux ? Ce n'est pas plus dur qu'un référendum

Merci

En cas de recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, comme le prévoit le présent projet de loi, le départ du personnel de la RATP sera décalé de 52 ans à 54 ans pour la catégorie B, c'est-à-dire les conducteurs,

Mais en supprimant ce régime avant toute négociation de branche globale aboutissant à une amélioration des conditions de travail, de salaires et de retraite de ces métiers,

pour laquelle l'ensemble des groupes de gauche et écologistes, mus par un devoir d'exemplarité et de cohérence, ont déposé une résolution invitant le bureau du Sénat à une réflexion transparente sur notre régime et sur son évolution, en lien avec le statut de l'élu.

avec les organisations syndicales et patronales, afin de favoriser l'attractivité des différents métiers et les déplacements de nos concitoyens et de nos invités. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

ne permet pas de disposer du temps nécessaire à la concertation avec les organisations syndicales et patronales représentatives. Je voterai

J'ai écouté attentivement l'intervention de M. Laménie, et je l'invite

proposez de monter les Français les uns contre les autres, en leur expliquant que, finalement, cela ne concernerait que quelques privilégiés et que tous ne seraient pas vraiment touchés. Vous essayez de créer de l'agitation à propos de soi-disant nantis parmi les travailleurs.

De manière cohérente, nous sommes fermement opposés à la suppression de l'ensemble des régimes spéciaux évoqués dans cet article 1, car nous considérons que ces mesures sont injustifiées. À ce titre, le régime spécial de retraite de la Banque de France est un exemple pertinent, puisqu'il est largement excédentaire, avec plus de 1,8 milliard d'euros reversés dans le pot commun depuis 2020. Ce régime spécial a donc une incidence positive certaine pour la préservation de notre modèle social. de notre modèle social. Il est excédentaire grâce à des surcotisations actées collectivement par les cotisants de ce régime. Les départs anticipés, à 57 ans notamment, ne concernent qu'une infime partie des agents, qui exercent les activités les plus pénibles. De plus, comme l'ont déjà rappelé certains de mes collègues, malgré le rôle central de la Banque de France, cette institution bicentenaire subit une diminution constante de ses effectifs et une dégradation continue des conditions de travail ainsi qu'une quasi-stagnation des salaires. Alors que le secteur privé possède déjà le quasi-monopole du secteur financier et bancaire, cette nouvelle attaque envers les agents de la Banque de France risque de profondément affecter le rôle joué par l'institution, que ce soit en matière de stratégie monétaire, de stabilité financière ou encore de services économiques rendus à la collectivité. Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, si votre objectif est de réaliser des économies, ne supprimez pas ce régime spécial, qui est excédentaire et qui participe du bon fonctionnement de cette institution.

en 2007, de la majoration de leur pension de retraite. Malgré les efforts consentis, le Gouvernement veut pénaliser encore ces agents. Le régime de retraite des salariés de la Banque de France s'autofinance grâce à des investissements. La caisse qui le gère peut verser 100 % des promesses de retraite faites aux agents. Ce régime s'équilibre de lui-même, entre les cotisations des agents- il comptait 7 850 cotisants en 2021 -, celles de l'employeur et les réserves accumulées pendant 215 ans.

en annonçant la fin de leur régime spécial par voie de presse, sans concertation préalable. Supprimer ce régime revient au fond à dire aux agents qu'ils auraient été gagnants à ne faire aucun effort. L'amendement

par démagogie, vous seriez mieux inspiré, monsieur le ministre, de retirer cette réforme et de reprendre de véritables négociations avec les partenaires sociaux, afin d'étudier, profession par profession, l'opportunité de revenir intégralement ou en partie sur certains régimes dits spéciaux. Une bonne réforme des retraites

de droite : « La Banque de France dispose d'une caisse de réserve des employés dont les capitaux sont placés. Cette caisse est alimentée par les cotisations des agents. La Banque se contente de verser si besoin un complément afin d'assurer l'équilibre financier du régime. Les promesses faites aux agents et aux retraités sont provisionnées à 100 % depuis 2019, avec des provisions comptables représentant 12 milliards d'euros en 2020. Cette façon de faire permet de distribuer des pensions essentiellement financées par les marchés financiers sans faire appel aux contribuables.

a été suivi d'un second, visant à la fermeture de quatorze caisses supplémentaires du fait de la diminution drastique de l'utilisation des espèces au quotidien par nos concitoyens.

La Banque de France rend des services d'intérêt général. Elle assure en effet une médiation du crédit, fournit des analyses de conjoncture et réalise des cotations économiques et financières d'entreprises, de collectivités territoriales ou de territoires. Pour les particuliers, elle gère les fichiers centraux de renseignements et traite notamment les cas de surendettement, ainsi que le droit au compte, qu'on appelle trivialement interdit bancaire. Les métiers de la Banque de France nécessitent de l'expertise de haut niveau, dans un contexte où les compétences financières sont très recherchées par des cabinets privés de cotation. L'attractivité du statut est un gage d'indépendance qui permet à la Banque de France d'assumer ses missions de service public dans de bonnes conditions.

Ce régime n'est pas le privilège de quelques-uns ; il s'inscrit dans le contrat national en matière de service public. Il n'y a donc absolument aucune raison de le supprimer.

C'est pourquoi nous nous opposons en tout point à la suppression des régimes spéciaux. L'urgence n'est pas là. Aujourd'hui, il faut protéger les Français qui sont en grande difficulté.

L'un des arguments du Gouvernement pour justifier la suppression de certains régimes spéciaux de retraite serait leur coût ; M. Dussopt l'évoquait tout à l'heure à propos de la RATP.

De plus, le régime spécial de la Banque de France ne correspond à aucun privilège, puisque les hommes et les femmes qui travaillent à la Banque de France partent à la retraite à 62 ans, comme le reste de la population et avec le même nombre d'annuités de cotisation.

J'observe que si l'on avait géré de la même manière la retraite des fonctionnaires, avec le même dispositif, la France aurait fait une économie budgétaire de l'ordre de 50 milliards comme il faut parfois faire un peu de politique, c'est un régime qui nous permet de constater ce qu'est une véritable conversion de la gauche. Jamais

défendre avec autant de vigueur un régime de capitalisation. Cher Pierre Laurent, vous avez eu des mots extraordinaires pour défendre la capitalisation,

au régime général des retraites, qui a été créé au lendemain de la guerre en 1945. Je veux rassurer mon collègue Étienne Blanc

à travers l'histoire un régime pionnier ou des régimes spéciaux, c'est bien parce qu'il existe parfois des spécificités qui doivent, tant sur le mode de financement que sur la reconnaissance de pénibilité, être

Mme la rapporteure générale

le régime de retraite de la Banque de France est bien un régime spécial. Il apparaît au neuvième alinéa de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, qui liste les régimes que l'on qualifie de « spéciaux

en cause : les excédents sont versés lorsque les produits des placements financiers qui sont l'actif du régime spécial de retraite permettent à la fois de couvrir l'intégralité des dépenses de pensions et d'apporter une participation sous forme de versement exceptionnel à l'État.

et si, pour une raison ou une autre, vous y travaillez moins de quinze ans, lorsque vous quittez l'établissement pour rejoindre un autre employeur, vous êtes reversé au régime général et vous perdez toute forme d'acquis au titre du régime spécial. En réalité, l'extinction à laquelle nous procédons permet aussi de rétablir une forme d'égalité, y compris parmi les actuels recrutés de la Banque de France. Enfin, je confirme les propos de Mme la rapporteure générale, et j'avais déjà souligné ce

et qui donnent satisfaction aux salariés comme d'ailleurs, dans un certain nombre de professions, aux hauts responsables et au patronat. Ces régimes, que ce soit celui des clercs de notaires ou celui de la Banque de France, sont très antérieurs à la création du régime général lors de la Libération. Or personne à l'époque n'a considéré nécessaire à l'égalité républicaine de mettre tout le monde sous la même toise.

Mais notre critique de la capitalisation est d'un autre ordre. Car ce que nous refusons, c'est le basculement de l'actuelle répartition vers la capitalisation. On peut avoir ce débat.

en l'occurrence, peu de valeur. Le gouverneur de la Banque de France, dont je pense qu'il doit savoir un peu compter, dit que ce régime ne correspond « à aucun privilège des hommes et des femmes de la Banque de France, qui partent à la retraite à 62 ans comme tout le monde, avec la même durée de cotisation La différence est qu'il « est provisionné dans nos comptes. C'est donc en réalité un régime autonome plutôt vertueux. » Ce régime est soutenu par les syndicats de la Banque de France et par le gouverneur de la Banque de France, et sa gestion est vertueuse. Deuxièmement,

par un régime lié à la situation particulière de la Banque de France, mais nous reconnaissons nous-mêmes depuis le début de ce débat qu'il peut parfaitement exister des régimes qui, fait de leur histoire, sont des régimes particuliers sans déroger aux règles générales. Mais puisqu'ils sont bien gérés, pourquoi les changer ? C'est exactement ce que nous disons. Allons au-delà des différences qui peuvent nous animer dans ces débats. Les groupes de gauche

parlementaires du groupe Les Républicains qui ont déposé un amendement identique. Si nous joignons nos voix et si tout le monde s'y met, nous aurons fait oeuvre utile cet après-midi en préservant ce régime.

Là encore, pourquoi vouloir démanteler un régime financièrement autonome ? Là encore, si ce régime spécial existe, c'est pour une raison bien particulière. Avant la mise en place de leur caisse, les salariés des études notariales n'avaient pas droit à une couverture de retraite, n'étant pas classés comme ouvriers ou fonctionnaires. Ils devaient pour ceux qui le pouvaient acheter des points de retraite auprès de la société de secours mutuel. Là encore, ce régime correspond à un souci de justice et de protection des salariés. Sa fermeture ne trouve donc aucune justification. La parole

Cela entraînerait de surcroît la fin de l'action sociale profitant aux salariés de la caisse. En contrepartie de cotisations supérieures à celles du régime général, les salariés du notariat bénéficient d'une pension de retraite

Pourquoi vouloir supprimer un régime qui est autosuffisant ? L'objectif est-il d'absorber les réserves de la caisse des clercs de notaires ? Interrogé par la profession, le Gouvernement n'a apporté aucune réponse. Silence ! Les débats à l'Assemblée nationale n'ont pas plus éclairé la situation. Afin de ne pas participer à une réduction drastique des droits à la retraite des clercs de notaire, nous nous opposons à la fermeture de leur régime spécial. La

pour objet la fermeture du régime spécial de retraite des notaires et clercs de notaire. Instituée par la loi du 12 juillet 1937, la caisse de retraite et de prévoyance des employés de notaire a représenté un véritable gain social pour les personnes réalisant des études notariales qui ne bénéficiaient logiquement pas encore d'un régime de retraite. Conservé lors de la création du régime général, ce régime spécial s'est progressivement développé en se concentrant uniquement sur les pensions de retraite. Comme cela a été rappelé, ce régime n'a jamais été déficitaire depuis sa création. En effet, grâce à une surcotisation importante des employés et à une contribution de 4 % des employeurs, ce régime est largement excédentaire et pérenne. Alors que la profession connaît déjà des difficultés pour recruter des personnels formés, une atteinte à son régime spécial pourrait fortement ralentir son développement. Il convient également de rappeler que l'âge de départ à la retraite pour ce régime est actuellement de 63 ans et dix mois. De plus, avec près de 88 % de femmes parmi les salariés du notariat, la suppression de ce régime porterait un nouveau coup dur à la retraite des femmes, qui subissent déjà une inégalité de salaire et des carrières souvent hachées. Ainsi, mes chers collègues, comme cela a été proposé sur plusieurs travées de cet hémicycle, revenons sur la fermeture de ce régime excédentaire et protecteur de ses salariés.

Il a strictement respecté les obligations diverses et variées qui ont pu lui être imposées au cours des réformes antérieures successives. Il est équilibré et juste pour tous les salariés du notariat. Cet équilibre a été obtenu par des efforts dont on ferait bien de s'inspirer, notamment en matière de ressources mobilisables pour le système de retraite : pas de plafond pour le calcul des cotisations ; prise en compte de la totalité des salaires et des primes dans l'assiette des cotisations. il existe bien d'autres pistes encore pour améliorer les recettes du régime de retraite, comme l'égalité salariale ou l'emploi des seniors. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans la suite des débats. l'amendement n° 669. Par cet amendement, nous souhaitons préserver le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaire. Ce régime compte 76 000 clercs et employés de notaire et 80 000 retraités. Instauré en 1937, le régime de sécurité sociale du secteur notarial a pour spécificité d'être doté de l'autonomie financière, d'être multibranches- maladie, retraite et recouvrement -et de servir une action sociale pour les personnes en situation de fragilité. Cette caisse est un régime excédentaire pérenne, financé par les cotisations supérieures des employés et abondé par la contribution de 4 % des employeurs, qui n'accorde

et néfaste pour son attractivité. Une étude de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications des collaborateurs du notariat indique qu'il manquerait 3 000 à 5 000 salariés

démagogique, il me semble que vous seriez mieux inspiré de retirer cette réforme, d'ouvrir de véritables négociations avec les partenaires sociaux et d'étudier, profession par profession, l'opportunité de revenir intégralement ou en partie sur certains régimes dits spéciaux. Une bonne réforme des retraites est une réforme qui allie sauvegarde de la répartition et progrès social ; ce n'est pas une réforme qui stigmatise certains et qui monte les Français les uns contre les autres. Les amendements

des actes de l'étude, des transactions immobilières, des successions et des donations. Surtout- et c'est peut-être le plus important -, ils vérifient l'authenticité des documents, des titres de propriété ou l'exactitude des inventaires. Ils transmettent, classent et répertorient tous les actes notariaux. Leur travail est assez stressant, dans la mesure où- on le sait très bien -les procédures notariales se sont considérablement complexifiées depuis quelques années. En outre, la dématérialisation, même si elle offre un réel confort aux signataires, est une source d'anxiété, d'angoisse pour ces clercs de notaire, qui sont chargés, souvent dans un domaine de compétence qui n'est pas le leur,

Bien au contraire, il a largement participé à la solidarité nationale en se faisant le vecteur de diverses compensations. Votre idéologie budgétaire tient donc là son antithèse. Mettre fin à ce régime financièrement autonome serait parfaitement injuste

Cette caisse, qui a été créée huit ans avant la sécurité sociale, n'avait aucune raison d'adhérer au régime général à la Libération. Pour autant, son autonomie n'a pas à être remise en cause aujourd'hui. à une bonne gestion, les clercs et employés de notaires ont créé un système excédentaire. Il serait donc profondément injuste de supprimer ce régime. À plusieurs reprises, les clercs ont prouvé leur capacité à se réformer.

Je voterai donc contre la suppression de ce régime.

car les clercs et employés de notaires sont confrontés à des conditions de travail particulières : horaires atypiques, rythme de travail soutenu, en plus de l'exigence de qualifications élevées.

des difficultés à l'avenir pour recruter et fidéliser un personnel qualifié, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité du service rendu aux usagers. C'est pourquoi nous sommes favorables au maintien de ce régime spécial. Avec cet amendement, nous proposons de préserver les droits et la protection sociale des clercs et des employés de notaires et, par la même occasion, la qualité du service rendu

Vous prenez la question à l'envers : plutôt que d'accorder des droits plus avantageux et, finalement, plus en phase avec la société à l'ensemble des salariés, vous préférez pénaliser celles et ceux qui bénéficient

pas la pénibilité, la souffrance au travail, l'usure et les difficultés. Longues études ou pas, longues carrières ou pas, tout le monde devra travailler plus longtemps. En fait, vous refusez absolument de voir cette logique selon laquelle il n'est pas

monsieur le ministre,

sécurité sociale. Je continue de ne pas comprendre pourquoi nous débattons de mesures qui n'ont pas d'impact financier sur le bilan rectificatif de la sécurité sociale. J'aimerais savoir ce que dit la note d'analyse du Conseil d'État sur le sujet

Les clercs de notaire, comme les notaires, pensent à l'avenir de leur métier et de leurs salariés. Franchement, monsieur le ministre, quand on voit les problèmes du pays, l'immense inflation, les graves difficultés de pouvoir d'achat, n'avez-vous vraiment rien d'autre à faire que de vous occuper des clercs de notaire, qui ne posent aucune difficulté à la Nation ? Je n'ai jamais entendu le matin en prenant mon café des gens me dire : « Madame la sénatrice, quel scandale ces clercs de notaire ! Ils sont en train de nous ruiner ! Quels privilégiés ! » Franchement, vous accumulez les mauvais coups, métier par métier, là où il n'y a aucune nécessité ! Nous voterons contre la suppression de ce régime.

Merci

Le scrutin est clos.

Le scrutin est ouvert.

Intervention après intervention, nous nous évertuons à démontrer l'intérêt plus que douteux de fermer les régimes spéciaux. À ce titre, l'exemple du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières est éclairant. Il est prévu de mettre un terme à ce régime, car il coûterait cher au contribuable. Or ce régime est à l'équilibre, grâce à la contribution tarifaire d'acheminement.

La fin du régime spécial entraînerait véritablement une perte d'activité, au moment où ce secteur connaît des difficultés de recrutement. Madame la rapporteure générale, vous avez évoqué l'évolution des métiers et la disparition,

... Ces emplois sont retenus dans le statut national du personnel des industries électriques et gazières pour relever du régime spécial de retraite. Ces métiers existent toujours. La pénibilité est toujours là. Comment les

a été supprimé. Faites les comptes et vous arriverez rapidement au résultat qui correspond au soi-disant déficit que nous sommes censés combler avec cette réforme ! Les superprofits, que vous refusez

vous voulez diviser les Français, mais ils comprennent que votre politique est de faire pleuvoir des milliards d'euros de cadeaux fiscaux sur les plus riches sur les plus grandes entreprises, qui accumulent comme jamais les profits depuis 2017. Voilà le fond du problème, et vous ne l'abordez jamais

Notre souveraineté énergétique commence par la souveraineté en compétences. La capacité de ces industries à recruter dépend bien sûr des salaires et des perspectives de carrière, mais n'oubliez pas que les conditions de retraite sont également un élément d'attractivité. Aussi,

Ce ne sont en aucun cas des privilèges ; ce sont des acquis- je dirais même que ce sont des conquis sociaux. La branche professionnelle des industries électriques et gazières regroupe 139 800 salariés et 160 employeurs. Ce sont les entreprises qui exercent en France des activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture d'électricité et de gaz, en particulier EDF et Engie, qui rassemblent 70 % des salariés de la branche. Ce sont ceux qui sont à pied d'oeuvre lorsqu'il y a une tempête ou des inondations, jusqu'à ce que le service public soit rétabli. Cela constitue des contraintes et des astreintes fortes. Dans ce secteur, les difficultés de recrutement sont nombreuses. Les entreprises doivent former des agents et des ingénieurs, que ce soit dans le nucléaire, l'hydraulique ou les énergies renouvelables. Elles s'efforcent de les garder et de les fidéliser,

En 2022, la caisse de retraite des industries électriques et gazières a rapporté 120 millions d'euros de plus que le versement des pensions au régime général. De plus, 1,6 milliard d'euros ont été versés au total entre 2005 et 2020 vers les régimes de retraite ayant moins d'actifs que de retraités, comme celui des agriculteurs ou des artisans. Ce régime ne coûte donc rien à la collectivité. Le supprimer ne rapportera aucune recette supplémentaire.

Ce statut a subi des attaques permanentes et, s'il comporte des avantages, c'est qu'il prévoit aussi beaucoup de servitudes, ainsi qu'un déroulement de carrière très modéré Ce régime spécial est la contrepartie de conditions de travail particulières et d'une forte pénibilité : astreintes, heures passées à genoux devant les coffres électriques, interventions exigeantes physiquement en haut des pylônes à toute heure du jour et de la nuit, Prendre en compte divers critères de pénibilité et les objectiver, c'est avant tout une mesure de justice sociale. Je le répète, ces régimes spéciaux sont la contrepartie de sujétions particulières. Cessons de niveler les droits des salariés par le bas, en supprimant les régimes spéciaux. Permettons au contraire que l'ensemble des salariés exposés à la pénibilité puissent partir plus tôt à la retraite. Par ailleurs, face aux défis

au dérèglement climatique qui a pour conséquence directe l'augmentation des événements météorologiques ayant un impact toujours plus fort sur les réseaux et que nous faisons face à une crise énergétique majeure du fait de la guerre en Ukraine, nous obligeant à réinterroger notre souveraineté énergétique. Supprimer brutalement les régimes dits « spéciaux » ne donne absolument aucun signe favorable envers ces secteurs pour des professions souvent très difficiles. Monsieur le ministre, plutôt que de tout supprimer de manière démagogique, il me semble que vous seriez mieux inspiré de retirer cette réforme, d'ouvrir de véritables négociations avec les partenaires sociaux et d'étudier, profession par profession, l'opportunité de revenir intégralement ou en partie sur certains régimes dits spéciaux. Une bonne réforme des retraites est une réforme qui allie sauvegarde de la répartition et progrès social ; ce n'est pas une réforme qui stigmatise certains et qui monte les Français les uns contre les autres. Les amendements

983. Le régime spécial des industries électriques et gazières concerne près de 140 000 salariés travaillant dans 157 entreprises de la branche.

est de 60 ans et devrait atteindre les 62 ans en 2024. Par ailleurs, revenir sur le régime spécial ne répond à aucune rationalité économique, puisque ce dernier est excédentaire. Cet excédent a d'ailleurs rapporté 120 millions

altérer considérablement cette confiance et compliquer la concertation. L'art de se tirer une balle dans le pied ! La seconde condition, c'est la capacité à mobiliser les compétences. Et là, on se tire une balle dans l'autre pied Le Gouvernement semble ne pas avoir compris que la situation énergétique de notre pays est extrêmement grave. Il s'agit d'un enjeu stratégique national de souveraineté, de compétitivité pour nos entreprises, de confort pour nos concitoyens et de décarbonation de notre économie dans un contexte d'urgence climatique. de décembre dernier indique que, pour construire de nouveaux réacteurs en France, la filière nucléaire doit recruter au moins 10 000 personnes par an à partir de 2023, dont 3 000 pour les seuls besoins d'EDF. Aucune filière industrielle n'a de tels plans de charge devant elle. Or que fait-on ? On réduit son attractivité ! Aussi, dans l'hypothèse où le régime spécial serait fermé, il est évident que, pour compenser ce manque d'attractivité, EDF devra offrir des augmentations salariales aux nouveaux entrants. Mais je ne pense pas

de notre modèle environnemental et de durabilité de nos politiques industrielles, singulièrement en matière de production énergétique. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait opportun de venir bousculer, par une réforme qui

Remettre en cause ces régimes spéciaux, c'est aussi diminuer l'attractivité des nombreux métiers des différentes filières concernées. Là encore, c'est une très grave erreur. Il est au contraire nécessaire de mettre en adéquation la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avec nos besoins. Nous avons voté récemment

du domaine de la loi ordinaire. De surcroît, les conséquences multiples de la suppression des régimes spéciaux qu'opère l'article 1 sont manifestes. Elles n'ont pas été évaluées dans toutes leurs implications productives, sociales et managériales, et leurs effets directs budgétaires ne sont pas avérés. Les futurs salariés des IEG n'ont pas à faire les frais des difficultés actuelles d'EDF, dont le seul responsable est l'État français, en particulier ceux qui l'ont dirigé depuis des décennies. La suppression des régimes spéciaux des IEG pour les seuls personnels recrutés à compter du 1 septembre 2023 est sans effet direct sur les dépenses et les recettes, puisqu'elle se borne à introduire un changement de régime d'affiliation de ces personnels au profit du régime général sans affecter directement le montant des cotisations versées. Elle n'a donc rien à faire dans un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. simplement que le grand oeuvre du président des riches et de ses gouvernements successifs est bien, depuis 2017, la suppression des statuts historiques qui ont contribué à la force industrielle et sociale de la France, telle qu'elle était issue du Conseil national de la Résistance. On savait que le ruissellement vers le bas était une fable. On voit ici que le ruissellement vers le haut est la nouvelle forme de spoliation de ce qui reste du capital social. Les Français l'ont compris, et ils vont vous le rappeler dans les jours à venir

plus vrai aujourd'hui que le mur des investissements dans les installations de production d'électricité est devant nous. La fermeture de ce régime spécial des métiers de l'énergie est un non-sens absolu, car ces métiers sont durs. Fermer ce régime est particulièrement brutal. Jusqu'à présent,

2007, on est passé à 43 ans. Or nous avons besoin de salariés qui se sentent bien dans leur travail ; c'est notre intérêt et c'est le leur. Nous avons tout simplement besoin de salariés de l'énergie et la question de l'attractivité se pose. La dureté du travail est évidente

pour rétablir l'énergie, par exemple lors d'une tempête, d'une inondation, d'un incendie ou d'une catastrophe industrielle, doivent être protégés. Nous avons bénéficié jusqu'à présent de leur travail et du service qu'ils nous ont rendu. nous avons toujours pu compter sur eux. Ils travaillent dans des environnements particulièrement extrêmes, par tous les temps, et je salue leur amour du bel ouvrage. Ils sont fiers de ce qu'ils font, et nous sommes satisfaits des services qu'ils rendent. C'est pourquoi ce régime spécial doit être maintenu.

À chaque fois, les élus et les ministres saluent ces agents et tirent une légitime fierté de ce service public qui sait se mobiliser pour rétablir des conditions de vie et de travail normales pour les Françaises et les Français. Ce régime spécial est mérité. Il vient saluer l'engagement et la pénibilité de ce travail. J'ai parlé des périodes exceptionnelles, mais je pourrais vous parler de de l'engagement de ces hommes et de ces femmes au quotidien : c'est moins spectaculaire, il n'y a pas de caméra de télévision, pas d'élu qui va à leur rencontre, mais, chaque fois qu'il y a un accident sur la route, qu'un camion rentre dans un pylône

la pénibilité du travail et l'engagement de ces hommes et de ces femmes au quotidien. l'amendement n° 1624. Cet amendement vise à ne pas fermer le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, qui s'applique aux 156 entreprises de la branche des IEG, dont EDF et Engie, et qui compte plus de 135 000 cotisants au 31 décembre 2021. EDF est le principal employeur du secteur, avec 44,7 % des effectifs des IEG. La réforme va supprimer les notions de service actif et de service insalubre, qui donnent droit à des majorations de durée permettant une retraite anticipée à ceux qui occupent ces postes pénibles. Le régime d'EDF prévoit une meilleure prise en compte de la pénibilité, car certains de ses travailleurs subissent une espérance de vie inférieure à la moyenne des Français ou des incapacités de travail importantes. Pour notre part, nous souhaitons que ces mesures protectrices, qui tiennent compte de la pénibilité des métiers, puissent être appliquées à l'ensemble des Français dont les conditions de travail sont pénibles et usantes.

combien les centrales nucléaires ont besoin de ces compétences ? Dès lors, pourquoi ne changeons-nous pas la politique énergétique en donnant un coup d'arrêt à ce que nous faisons depuis vingt-cinq ans dans ce domaine et en refusant de passer au régime général ?

Monsieur le ministre, pour reprendre une expression maintenant consacrée par l'un de vos collègues, vous avez donc décidé de « bordéliser » un secteur majeur de notre souveraineté énergétique C'est un choix extrêmement lourd, et les mobilisations ont commencé dès aujourd'hui chez ces personnels, qui ont été décrits avec beaucoup de force, de vigueur, de justice et de justesse par nos collègues. Ce régime de retraite ne date pas d'hier : il a été fondé en 1859 par les salariés de la compagnie parisienne du gaz à partir d'une caisse de secours et de prévoyance- d'autres entreprises ont ainsi pu créer leur régime. Au moment de la création du régime général des assurances sociales en 1930, puis en 1945, certains travailleurs bénéficiant de régimes de retraite plus protecteurs ont été reconnus.

le régime de retraite des IEG symbolise finalement une période chère à notre coeur à toutes et tous, celle du Conseil national de la Résistance

Et j'ai dit ce matin que vous raisonniez à l'inverse, en pensant que la suppression des régimes spéciaux allait aplanir les conflits d'identité dans notre société : je crains, au contraire, qu'elle ne les exacerbe. En fait,

ne marche pas ainsi dans la vie. Leur savoir-faire, leur expérience, leur stabilité ne font pas d'eux des êtres totalement adaptés en permanence aux besoins du marché. En fait, en vous attaquant aux régimes spéciaux, vous dévalorisez l'identité, le savoir-faire la fierté que donnent un métier et l'appartenance à une entreprise aussi importante dans le service public des Français que celle qui fait l'objet de cet amendement. L'amendement présenter l'amendement n° 2261. Mes chers collègues, en vous entendant, depuis ce matin, sur la suppression des régimes spéciaux, je me dis que nous ne devons pas être nombreux à avoir des parents ayant exercé des métiers pénibles.

Vous demandez aujourd'hui la suppression de leurs régimes spéciaux, qui est une mesure de justice sociale et d'équité prenant en compte la pénibilité de leur travail. Chers collègues, auriez-vous la mémoire courte ?

Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes, de ces personnels qui sont aujourd'hui un enjeu stratégique pour notre pays. Enfin, le régime de retraite des industries gazières et électriques est adossé au régime général depuis 2008. Il ne doit rien à la solidarité nationale ; au contraire, il y contribue, en lui apportant des recettes. Au travers du slogan « on meurt plus tôt, on part plus tôt », ce régime est présenté comme un régime pionnier par ses bénéficiaires, prenant en compte la pénibilité au travail liée à une espérance de vie entamée et au bouleversement des conditions de vie. Mes chers collègues, leur régime si spécial doit être maintenu. Je vous le demande

tributaire ni de l'État ni des autres régimes. Pourquoi cet acharnement à le supprimer ? Pour des raisons financières ? Non, car le régime est excédentaire. Pour des raisons d'équité ? le régime participe au financement d'autres régimes, qui comptent moins d'actifs que de retraités, comme ceux des agriculteurs et des artisans. En raison de la contribution tarifaire d'acheminement, censée coûter 1,7 milliard d'euros aux usagers ? Pourtant, cette contribution est une imposition de toute nature, et non une aide d'État qui se substitue- c'est le choix qui a été fait lors de la libéralisation du secteur en 2004 par le gouvernement Raffarin -à la part du tarif d'électricité et de gaz naturel, qui a assuré son financement, la part des droits spécifiques passés correspondant aux activités régulées. La CTA est acquittée sur le prix global par le client final, donc par le contribuable. Comment pouvez-vous garantir la pérennité du régime, alors que nous savons que la fameuse clause du grand-père conduira à appliquer le régime général à tout nouvel entrant, avec par conséquent de moins en de moins en moins de cotisants ? Ce régime ne pourra pas survivre. Aucune des raisons que vous invoquez ne tient donc la route. Ne nous y trompons pas : aujourd'hui comme en 2004, la suppression du régime des IEG est à chercher dans votre volonté de démantèlement du service énergétique français, c'est-à-dire dans dépeçage et de dislocation d'EDF un plan Hercule qui peut revenir à chaque instant, malgré l'opposition unanime des organisations syndicales et de ceux qui défendent un service 100 % public. Engie, entreprise privée, n'a jamais caché son rêve de sortir du statut national. C'est la seule justification de l'article 1, que ce soit pour les IEG ou la RATP. L'amendement Le régime des électriciens et gaziers est profondément lié à l'importance que notre pays accordait à la question énergétique et à la volonté de bâtir des entreprises publiques puissantes, capables de relever les défis de l'électrification de notre pays de l'après-guerre. Ce régime s'est consolidé au fil du temps pour garantir aux électriciens et aux gaziers un haut niveau de droits, correspondant aux contraintes et à la pénibilité de leur mission. On parle ici de femmes et d'hommes profondément engagés dans le service public de l'électricité et du gaz. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau face à des défis majeurs : relance du nucléaire en France, construction de nouveaux EPR, nécessité de renforcer nos réseaux de distribution pour faire face à l'essor des énergies renouvelables, déploiement au niveau industriel du véhicule électrique ... La liste est loin d'être exhaustive. Pour assurer cette transition énergétique, il faudra des agents de plus en plus qualifiés. Il sera nécessaire de consolider les compétences et les savoir-faire et de recréer un tissu industriel de qualité. En effet, aujourd'hui, le régime spécial de retraite des IEG fait partie d'un pacte global, qui reflète notamment un certain nombre d'astreintes et de difficultés au travail. Dès lors, quelle erreur historique que de vouloir supprimer un régime qui est aussi un vecteur d'attractivité dans un secteur essentiel ! La suppression du régime spécial des IEG ne traduit, en vérité, que votre volonté de remettre en cause leur statut et d'achever, par là même, les missions de service public.

Les électriciens et les gaziers cotisent à un niveau supérieur et se constituent mutuellement des droits à la retraite correspondant à leur situation. C'est un modèle vers lequel il faut se tourner. Il s'agit, à nos yeux, non pas de régimes spéciaux, mais, je le réaffirme, de régimes pionniers. Nous sommes attachés à la défense de ces conquis sociaux. C'est pourquoi nous demandons la suppression la suppression des alinéas 15 et 16. effet, nous discutons non pas d'un régime de retraite, mais du pacte que nous allons passer pour l'avenir, ou que nous allons rompre, avec l'ensemble des salariés des industries électriques et gazières. Nous savons tous que la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays est de nouveau une question d'avenir et qu'elle est sur la table. Il va falloir procéder à la plus grande mutation de notre système électrique depuis la construction du parc électronucléaire et du parc hydraulique de la France. France. Soit nous sommes capables de réussir cette mutation, et nous répondrons possiblement aux enjeux d'industrialisation, de souveraineté et d'urgence climatique, avec du nucléaire et avec des EnR, soit nous n'en sommes pas capables, et alors rien ne sera possible. Or nous n'y parviendrons pas sans une mobilisation générale et durable de l'ensemble des professions IEG dans le pays. Votre projet fait exactement l'inverse il propose, au travers de cette question de régime de retraite, de rompre le pacte national qui a été passé avec les salariés des IEG depuis la Libération.

tout le pays -, pour s'opposer au projet que vous voulez passer en force. Ce pacte, vous l'avez déjà beaucoup abîmé. La question qui est devant nous est de savoir si vous allez l'achever ou si, au contraire, nous allons le relancer pour l'étendre à toutes les professions IEG d'aujourd'hui et à celles que nous devrons embaucher et former pour construire la réussite du nouveau projet énergétique pour la France.

sur les régimes spéciaux, notamment sur celui des gaziers. C'est pourquoi nous avions décliné un certain nombre d'amendements, visant

Je veux aussi associer à cet hommage tous ceux qui interviennent pour la maintenance du réseau et qui sont des sous-traitants. De fait, 80 % de travaux de maintenance sont réalisés par des sous-traitants qui, eux, n'ont pas de régime spécial

Monsieur le ministre,

que, demain, l'ensemble des salariés des IEG seraient privés de leur régime spécial ne sont pas dans le vrai. Ce sont uniquement les nouveaux qui le seront. Cela m'amène à un point qui a été évoqué rapidement, à savoir les conséquences de ce que l'on pourrait appeler le « tarissement du flux », par rapport à un régime spécial qui doit gérer les retraités actuels et celles et ceux qui gagneront leur retraite sous couvert, toujours, de ce régime. Nous l'avons déjà fait pour la SNCF, lorsque nous avons mis en place l'extinction du statut- et pas seulement, pour le coup, du régime d'assurance vieillesse.

qu'il n'y a pas d'excédent. Il peut y avoir parfois, telle ou telle année, des reversements. Mais un régime qui s'équilibre et qui produit de légers excédents

Vous avez parlé, dans une intervention précédente, de « situation de rente ». Quelle blague ! Les vraies situations de rente sont pour celles et ceux qui profitent de la crise et que vous exonérez systématiquement de toute contribution et de toute

Ils ont bien conscience que votre politique ne va toujours que dans un seul sens. Cette brutalité suscite la colère légitime de nos compatriotes, qui manifestent en masse pacifiquement depuis plusieurs semaines, dans une situation économique pourtant très difficile, où ils doivent la plupart du temps se priver de journées de salaire pour défendre un droit collectif, celui de bénéficier, après une vie de travail, d'une pension de retraite décente à un âge décent.

Pendant longtemps, les Français ont été fiers de leurs services publics de l'électricité et du gaz, de la SNCF, de leurs hôpitaux et de leur école publique. étaient fiers du modèle républicain, cette sorte d'armature qui servait aussi au développement économique du pays. Or ils constatent que vos choix libéraux ont détricoté et affaibli considérablement ces piliers de notre République et de notre pays. Et vous nous donniez des leçons :

vraiment la preuve -, qui reposent sur la pleine mobilisation des salariés dans l'exercice de leur mission de service public, s'apparente davantage à de la provocation qu'à une quelconque volonté de justice entre les salariés du régime général et ceux des services publics.

Combien de personnes seraient concernées ? Surtout, sont-elles véritablement trop avantagées ? Seraient-elles des nantis ? Monsieur le ministre, permettez-moi une petite incursion dans ma vie privée. Il se trouve que je suis la fille d'un gazier qui est aujourd'hui à la retraite. Or je ne crois pas qu'il ait été un nanti, un privilégié. Il a exercé ses missions, ses fonctions, son métier dans les conditions qui étaient les siennes, parfois difficiles, et, comme cela a été dit par mes collègues, parfois, aussi, au péril de sa vie. Mais il fallait exercer cette mission de service public ! Alors, non, il n'y a pas de nantis ! Il n'y a pas de privilégiés. Enfin, à vous écouter, monsieur le ministre,

Dans l'étude d'impact, il est précisé que la suppression devrait conduire à ce qu'il y ait 4 490 nouveaux affiliés au régime général entre septembre et décembre 2023, et autant de moins pour les régimes concernés, qui

pas au banc du Gouvernement ! Ils sont dans la rue, pas aux côtés de ceux qui mettent en pièces le régime de sécurité sociale des agents d'EDF

d'agents, hommes et femmes, gaziers et électriciens qui, depuis 1946, sont l'honneur industriel de la France.

de vente à la découpe d'EDF et de ce qui reste de Gaz de France. Cette idée n'a jamais quitté l'esprit des gouvernants actuels.

Ces régimes ont toujours contribué à la solidarité nationale, en reversant leurs excédents aux caisses déficitaires. Par ailleurs, je rappelle que ces salariés que vous pointez du doigt cotisent à hauteur de 13

Vous avez déclaré que ce régime pesait 1,7 milliard d'euros. Or vous avez fait cadeau de centaines de milliards d'euros aux grands patrons sans aucune contrepartie- cherchez l'erreur

il est impensable de faire cohabiter deux régimes. Outre l'injustice pour les nouveaux embauchés, qui devront accomplir les mêmes tâches que leurs collègues, mais en relevant d'un régime différent, ces travailleurs et travailleuses savent bien qu'il s'agit de la disparition assurée et assumée de leur statut. Comment pouvez-vous nier la dégradation rapide de l'équilibre entre cotisants actifs et retraités, qui constituera un énième prétexte pour remettre en cause les dispositifs statutaires ? Or ce statut et ces régimes spéciaux de retraite et et gazières (Camieg) -sont la juste contribution sociale due aux agents qui assurent le service public de l'énergie 365 jours par an et 24 heures sur 24, et par tous les temps, pour la Nation et les usagers.

Monsieur le ministre,

Le scrutin est clos.